La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 9 décembre 2021 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. L'ordre du jour appelle les réponses à des questions orales.

et à la manifestation de la vérité. Contrairement aux idées reçues, la médecine légale s'occupe minoritairement des personnes décédées et majoritairement des personnes vivantes. Parmi elles figurent notamment les femmes victimes de violences intrafamiliales. En tant que présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances Le Gouvernement y attache également un grand intérêt, puisque, en déclarant l'égalité entre les femmes et les hommes grande cause du quinquennat, en décrétant que l'accompagnement des victimes constituait l'un des trois piliers de cette grande cause en souhaitant permettre le recueil de preuves sans dépôt de plainte dans les unités médico-judiciaires, il a conféré aux médecins légistes une mission essentielle. En Vendée, le faible effectif de médecins légistes, qui représente actuellement 0,8 équivalent temps plein (ETP), ne permet pas une prise en charge médico-légale

En conséquence, cette charge incombe à des professionnels de santé déjà sous tension, urgentistes et médecins généralistes, qui ne disposent pas forcément des compétences requises par l'exercice de la médecine légale. Le département voisin de la Charente-Maritime, qui présente des caractéristiques semblables à la Vendée, a obtenu la validation d'un projet de service de médecine légale adulte et compte désormais 6,2 ETP. Bien qu'elle ait présenté un même projet, la Vendée ne peut y prétendre.

Aux termes du schéma directeur de la médecine légale résultant des circulaires des 27 décembre 2010 et 25 avril 2012, la thanatologie dans le département de la Vendée, soit sur le ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne, relève du centre hospitalier universitaire de Nantes. La médecine légale du vivant relève quant à elle du réseau de proximité, qu'il s'agisse des médecins libéraux, des urgences ou des associations de médecins. Dans le cadre de la justice de proximité, j'ai obtenu la somme de 20 millions d'euros pour la médecine légale du vivant. Le déploiement de ces fonds vise au renforcement des structures locales, sans modification du schéma directeur. À cette fin, un recensement des besoins a été réalisé sur la base d'une évaluation chiffrée de l'activité des différents ressorts. Si les ressorts des tribunaux de Poitiers de Poitiers et de La Rochelle ont été identifiés dans ce cadre, la situation de la médecine légale dans les ressorts de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne, à l'heure où je vous parle, n'a pas été identifiée comme se trouvant en difficulté, les données d'activité y étant bien inférieures à celles du département de la Charente-Maritime. Interrogée dans ce cadre, la cour d'appel de Poitiers n'a pas évoqué la situation de la médecine légale dans le département de la Vendée comme posant problème. Ce ressort pourra néanmoins faire l'objet d'une nouvelle analyse dans le cadre de la réévaluation globale des moyens qui aura lieu en début d'année 2022.

En effet, cette promiscuité entraîne d'importantes tensions entre les détenus eux-mêmes, et avec les surveillants. Les incidents se multiplient depuis plusieurs années sans qu'aucune solution soit apportée À cela s'ajoutent des contraintes supplémentaires liées d'une part à la crise sanitaire, qui conduit à l'isolement systématique des nouveaux détenus pendant sept jours, et, d'autre part, aux travaux de rénovation qui demanderont de libérer des cellules. Pour rappel, le Gouvernement avait renoncé en 2018 au projet de construction d'une nouvelle prison en Vendée. À la suite de cette annonce, la garde des sceaux s'était engagée à débloquer 4 millions d'euros pour rénover les prisons vendéennes. Ces travaux, quoiqu'ils soient nécessaires, n'amélioreront malheureusement pas la situation de surpopulation carcérale. En avril dernier, le Premier ministre a annoncé un plan « 15 000 places de prison ». Or aucune nouvelle place n'est prévue en Vendée, alors que les deux prisons de notre département présentent un taux de surpopulation carcérale parmi les plus élevés de France.

Or la direction interrégionale des services pénitentiaires Grand-Ouest est particulièrement marquée par la surpopulation et le sera davantage à l'avenir. Le choix a donc été de prévoir la création de deux établissements pénitentiaires à Vannes, pour 550 places, et à Angers, pour 850 places. L'engagement du Gouvernement s'est aussi largement porté sur la nécessité d'assurer la maintenance et la rénovation des établissements existants, moyen, je le rappelle, d'un budget de 138 millions d'euros pour 2022, contre 60 à 80 millions d'euros consacrés annuellement à ces postes entre 2014 et 2016. Dans votre département, une somme de 4 millions d'euros a été budgétée pour rénover les maisons d'arrêt. Il s'agit cependant d'un exercice complexe, qui nécessite le transfert d'une partie des détenus d'une structure vers une autre, ce qui a un impact sur la programmation des travaux.

Avec une maternité de moins, le centre hospitalier de Montauban et la clinique Boyé connaîtront un regain d'activité très important, qu'il sera possible d'absorber dans un premier temps, mais dans un premier temps seulement, car la dynamique démographique de mon département est particulièrement forte. De plus, avec seulement deux maternités, c'est tout simplement le libre choix de son lieu d'accouchement qui se trouvera limité. de l'autonomie, trouvez-vous normal que le groupe Elsan puisse décider unilatéralement de cette fermeture ? Surtout, que compte faire le Gouvernement pour garantir à l'avenir une offre suffisante pour les futures mères de Tarn-et-Garonne ? La parole

Cette préoccupation est partagée par le Gouvernement. Dans le cas présent, comme vous le rappelez par ailleurs, cette fermeture n'est nullement réalisée sur l'initiative des pouvoirs publics, mais résulte d'une décision de gestion d'un groupe privé de cliniques. L'ARS Occitanie et sa délégation départementale de Tam-et-Garonne ont suivi de près ce dossier en organisant des réunions régulières associant les directeurs des trois établissements porteurs de maternité dans le département, pour préparer la transition. Depuis l'annonce de cette fermeture, les femmes qui souhaitaient accoucher à la clinique du Pont de Chaume sont progressivement accueillies au centre hospitalier de Montauban et à la clinique Boyé. Notre priorité est de nous assurer que ces prises en charge s'effectuent dans les meilleures conditions de sécurité, mais aussi de respect du libre choix des femmes. La délégation départementale accompagne, avec l'appui du réseau de périnatalité Occitanie, les sages-femmes et les gynécologues-obstétriciens pour consolider la filière périnatalité et sécuriser l'offre de soins dans le département. Enfin, comme vous le soulignez, la clinique du Pont de Chaume a bien perçu une aide financière dans le cadre des investissements du quotidien des établissements de santé. Il ne s'agit pas là d'un financement pour un projet de transformation du bâti.

La Caisse des dépôts et consignations s'assure par ailleurs de l'adéquation entre l'objet contractualisé et les factures présentées. Aucun soutien financier ne sera donc apporté pour des engagements non tenus.

au niveau tant humain qu'économique, et l'importance des dégâts qu'elle a causés est encore sous-estimée. En effet, outre les formes graves et immédiates d'infection au SARS-CoV-2, qui nécessitent des soins hospitaliers importants et entraînent une prise en charge à 100 % la reconnaissance d'une affection de longue durée, ou ALD, une autre forme de covid-19 affecte les patients à plus long terme : le covid long. D'après les informations de la Haute Autorité de santé, concerne plus de 20 % des personnes ayant contracté le coronavirus. Il touche des patients ayant présenté une forme bénigne de la maladie dans un premier temps, mais qui subissent de lourds symptômes à long terme troubles cardiaques et/ou respiratoires, fatigue intense, pertes de mémoire, etc. Cela peut aller jusqu'à affecter leur capacité à travailler, avec les conséquences dramatiques que cela implique. Les médecins s'accordent à dire que, pour soigner cette forme de covid-19, il est nécessaire d'accéder à une prise en charge rapide et pluridisciplinaire : neurologique, cardiaque, pulmonaire, musculaire et psychologique. Or nombreux sont les patients qui voient leur demande d'ALD refusée par la caisse primaire d'assurance maladie, au motif qu'ils n'entrent pas dans l'une des trois situations justifiant la prise en charge. Pendant ce temps, aux États-Unis, le président Biden reconnaît le covid long comme une forme de handicap, et le Royaume-Uni a mis en place une nomenclature adéquate pour permettre sa prise en charge.

Madame la sénatrice Michelle Gréaume, vous appelez mon attention sur le besoin exprimé d'une prise en charge pluridisciplinaire du covid long à 100 %. La prise en charge des patients souffrant de troubles persistants de la covid-19 constitue l'une de nos priorités, que nous sommes en train d'analyser. Tout d'abord, on distingue les patients souffrant de symptômes persistants pendant quatre à douze semaines, que l'on qualifie de « covid long

difficile à évaluer, puisque les troubles peuvent aller de la simple anosmie à une perte d'autonomie invalidante. Ayant écouté les recommandations de la HAS, le ministère des solidarités et de la santé a souhaité organiser l'offre de soins, afin d'assurer une prise en charge pluridisciplinaire aux patients. Cette prise en charge s'articule autour du médecin traitant traitant chargé du repérage, d'éventuelles consultations spécialisées, selon les symptômes, et d'une prise en charge en soins de suite et de réadaptation pour les cas les plus sévères. Des cellules de coordination post-covid ont été mises en place sur l'ensemble du territoire. Elles ont pour objectif d'orienter, d'accompagner et de coordonner les patients et les professionnels.

la diversité des symptômes ne permettent pas d'envisager la création d'une ALD spécifique, faute de définition et de critères précis. Néanmoins, certains patients sont déjà admis en ALD, soit dans le cadre d'une

le préjudice est lourd pour les malades et touche plusieurs domaines : financier, médical, psychologique. Des patients franchissent les frontières pour tester des traitements aussi onéreux que hasardeux, sans certitude quant à leur efficacité, en désespoir de cause et faute de trouver une réponse à leurs maux en France. Enfin, une sensibilisation large doit être réalisée. Les nouvelles fiches de suivi de la Haute Autorité de santé sont en ligne, sans écho dans l'espace médiatique. Ces fiches doivent être diffusées largement, dans chaque cabinet médical, et dans tous les centres de prise en charge. La parole est à Mme Sylviane Noël,

des maires déplorent la multiplication des déserts médicaux. Les situations de ce type se comptent par milliers, laissant des malades et des familles entières en pleine détresse. Si les causes de ces tensions sont nombreuses et anciennes, le surmenage des personnels et, surtout, l'obligation vaccinale des soignants ont été la goutte de trop. Alors qu'il y a dix-huit mois les soignants assuraient sans sourciller leur activité, sans masque, sans blouse, sans gants, sans gel, priés de venir travailler même s'ils étaient atteints du covid-19, ces mêmes personnels se trouvent aujourd'hui démis de leurs fonctions, sans revenus, sans statut, sans aucune considération s'ils choisissent d'exercer, comme tous les autres citoyens de notre pays, leur libre choix à l'égard de ce vaccin. Les héros d'hier sont les parias d'aujourd'hui ! Il y aurait ainsi 15 000 soignants suspendus en France : 15 000 personnes de perdues pour les établissements de santé et plongées dans la précarité.

Madame la sénatrice Sylviane Noël, au travers de votre question, ce que vous demandez, c'est que le Gouvernement revienne sur le principe de l'obligation vaccinale des soignants dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux, comme si cette décision était à l'origine du désengagement soudain des établissements.

94 % des salariés et agents justifiaient d'un schéma vaccinal complet et moins de 0,6 % des professionnels concernés par l'obligation vaccinale avaient fait l'objet d'une suspension- soit une personne pour deux cents Les dernières enquêtes ont montré que bon nombre de suspensions étaient levées progressivement et que, dans deux situations sur trois, la levée de suspension était liée à l'adhésion à l'obligation vaccinale. Non, madame la sénatrice, « les héros d'hier ne sont pas les « parias d'aujourd'hui », bien au contraire. Les soignants continuent de faire preuve d'un engagement remarquable. Ils ont adhéré massivement à l'obligation vaccinale, par déontologie, par devoir, pour protéger leurs patients et les plus fragiles. Les soignants qui n'ont pas encore adhéré à l'obligation vaccinale ne sont pas des personnes perdues. Ce sont des personnes qui ont encore le choix et qui peuvent dialoguer avec leur établissement. Cependant, les réadmettre dans les établissements reviendrait à exposer les patients à un risque plus élevé de contamination. Nous ne pouvons pas l'accepter, évidemment, surtout dans le contexte actuel de cinquième vague. Le principe de l'obligation vaccinale doit donc être

Combien d'enfants ne sont-ils pas pris en charge par des unités pédopsychiatriques complètement saturées ? Face à cette situation, le Gouvernement préfère renvoyer des personnels dans un moment de très forte tension hospitalière,

soit un différentiel entre les annonces et les versements attendus de la part de l'État de 75 % pour les unités de soins de longue durée, 30 % pour les Ehpad, 20 % pour les services de psychiatrie et 18 % pour les soins de suite et de réadaptation. Cette situation est inacceptable, car elle exerce une pression intolérable sur les établissements placés auprès des personnes fragiles, alors que la cinquième vague de covid-19 est déjà là et que ces professionnels ont toujours répondu présent. Je vous demande de vous engager au versement des aides annoncées avant la fin de l'année, faute de quoi ces structures seront en grande difficulté, alors qu'elles espéraient participer de la juste et nécessaire revalorisation de leurs salariés promise par le Gouvernement. Ôtez-moi d'un doute, n'y aurait-il plus assez de sous dans les caisses du ministère ? ... Par

d'allocation des crédits. Les financements restants seront délégués par la troisième circulaire de campagne de fin d'année. Si l'accord du Ségur visait prioritairement les soignants de structures publiques, le Premier ministre a annoncé une revalorisation des médecins des hôpitaux privés non lucratifs. En outre, dès juillet 2020, la transposition du Ségur a été prévue pour les personnels non médicaux.

le bénéfice de la mesure socle aux personnels soignants, auxiliaires de vie sociale, aides médico-psychologiques ou accompagnants éducatifs et sociaux exerçant dans les accueils de jour autonomes et dans les résidences autonomie. L'ensemble de ces mesures entrera en vigueur au 1 novembre 2021 dans le secteur privé non lucratif. Enfin, le Premier ministre a annoncé, pour 2022, une conférence des métiers de l'accompagnement social et médico-social, qui permettra de fixer le cap et la méthode,

Outre les préoccupations des ménages en matière de coût de l'énergie et des carburants, plusieurs millions de nos concitoyens souffrent encore de la faim. Le constat est alarmant la direction générale de la cohésion sociale estime qu'entre 5 et 7 millions de Français ont eu recours à l'aide alimentaire en 2020, contre 5,5 millions en 2017 et 2,6 millions en 2006. Les confinements et la crise sanitaire ont, certes, provoqué un choc budgétaire supplémentaire chez les familles les plus pauvres ; pourtant, c'est la tendance mesurée sur le temps long qui doit nous alerter, soit une insécurité alimentaire qui toucherait près de 10 % de la population. Loin de ne concerner que les sans-abri ou les étrangers en situation irrégulière, le besoin d'aide alimentaire est aussi massivement exprimé par des travailleurs, des retraités et des étudiants. On ne saurait ignorer ni leur détresse sociale ni les risques sanitaires qui pèsent sur eux. À ces tristes observations s'ajoute le fait que l'aide alimentaire repose essentiellement sur la redistribution de produits invendus. Comment se satisfaire, dans un pays reconnu pour sa gastronomie et la qualité de ses productions agricoles, de ne céder aux plus vulnérables d'entre nous que les « restes » d'une société surconsommatrice, rendue malade par ses inégalités ? Aucune « indemnité inflation », aucun semblable expédient palliatif ne saurait soulager durablement ces milliers de familles éprouvées par la précarité alimentaire. Aussi ma question est-elle simple : quelles mesures le Gouvernement entend-il prendre pour faire advenir les conditions d'un accès digne,

accompagnent les collectivités territoriales dans la gestion de leur personnel en ce qui concerne la santé et les conditions de travail ; pour cela, ils disposent d'un service de médecine préventive, afin de renforcer et de compléter l'action du service hygiène et sécurité. Leur mission est d'éviter toute altération de l'état de santé des agents en raison de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène, les risques de contagion et l'état de santé. En cette période de pandémie, durant laquelle les salariés sont fragilisés, leur rôle est d'autant plus important qu'ils participent à la lutte contre la propagation du virus. Pour assurer leur mission, Pour assurer leur mission, les centres de gestion doivent recruter des médecins ayant la qualification « santé au travail ». Malheureusement, peu de médecins la détiennent. En revanche, nombre de facultés de médecine, notamment celle de Reims, ou d'institut en médecine agricole, comme celui de Tours, délivrent des diplômes universitaires portant cette mention. En Seine-et-Marne, le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CDG77) ne parvient pas à obtenir de réponse claire sur la valeur de ces diplômes ou de ces titres pour exercer dans les services de médecine préventive des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. La reconnaissance de ces titres obtenus par des médecins généralistes en exercice, souhaitant bien souvent une reconversion et ayant suivi deux ans d'études, aiderait grand nombre de centres de gestion, voire de collectivités territoriales. Une information précise permettrait de lever les interrogations qui subsistent sur ces recrutements. Si l'équivalence de ces diplômes universitaires devait être reconnue, sera-t-elle acquise pour l'ensemble de leur carrière, comme une sorte de validation des acquis de l'expérience ?

déléguée chargée de l'autonomie. Madame la sénatrice Colette Mélot, les conditions d'exercice de la médecine préventive, garantes de la qualité des soins, sont définies par voie réglementaire. Pour exercer la médecine préventive, les médecins doivent être qualifiés en médecine du travail ou en médecine et santé au travail, spécialité créée depuis la réforme du troisième cycle des études de médecine de 2017. Ils peuvent également être titulaires d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels. C'est la réponse pour l'immense majorité des cas. Pour autant, la reconnaissance de la qualification peut s'appuyer sur d'autres leviers. Ainsi, la détention d'un diplôme universitaire portant la mention « santé au travail » peut être un argument pour faire valoir une reconnaissance de qualification en médecine et santé au travail auprès de l'Ordre des médecins. Cependant, ce diplôme seul ne pourrait suffire à permettre aux médecins qualifiés en médecine générale l'exercice au sein des centres de gestion que vous mentionnez. Dans cette situation, la qualification est donc appréciée au cas par cas par les autorités compétentes. Vous m'interrogez également sur l'accès à cette discipline de médecins ayant obtenu des diplômes étrangers. Comme vous le savez, pour exercer la médecine en France, tout titulaire d'un diplôme autorisant l'exercice de la médecine obtenu dans d'autres États autres que les États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou encore que ceux avec lesquels un accord bilatéral existe, doit nécessairement obtenir une autorisation pour l'exercice en France, délivrée par le Centre national de gestion. Il n'est donc pas permis aux établissements de procéder à des recrutements de gré à gré. En l'espèce, un praticien titulaire d'un diplôme délivré par l'Algérie ou le Maroc pourra ainsi être autorisé à exercer sa spécialité en France, après avoir, d'une part, d'une part, satisfait aux épreuves de vérification des connaissances (EVC) organisées chaque année par profession et par spécialité, et, d'autre part, accompli un parcours de consolidation des compétences d'une durée de deux ans au sein d'un des postes arrêtés chaque année. Il s'agit d'une condition essentielle pour assurer que les prétendants disposent de l'ensemble des compétences attendues pour l'exercice dans ces spécialités. La

particulièrement inquiétante ces derniers mois sur le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque, particulièrement dans la commune de Cappelle-la-Grande. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : de 2010 à 2020, dans la communauté urbaine de Dunkerque, le nombre de médecins généralistes est passé de 220 à 163. Près de 40 % de ces médecins ont plus de 60 ans et partiront donc à la retraite dans les prochaines années. Ces chiffres doivent d'ailleurs être croisés avec la démographie de la population senior, laquelle ne cesse d'augmenter sur ce territoire. Cappelle-la-Grande, commune de près de 8 000 habitants, passe de 10 médecins présents en 2010 à 1 seul en 2022, âgé, qui plus est, de 71 ans. La commune s'est retroussé les manches afin d'endiguer cette situation, malheureusement en vain, malgré des possibilités d'accompagnement et la mise à disposition de locaux. De nombreux territoires en France, en zones rurales ou en quartiers prioritaires, sont confrontés à la même situation. Pour autant, dans le département du Nord, l'accès à la santé doit être, plus que jamais, une priorité, puisque, à tous les âges, les indicateurs de santé sont au rouge. Sans accès à un médecin de proximité de confiance, le parcours de santé peut se dégrader très vite. Pour faire face au problème des zones dénuées de médecin, un certain nombre de collectivités ont fait le choix d'être à l'initiative. Ainsi, le département du Pas-de-Calais vient d'annoncer récemment le choix d'expérimenter sur trois ans le recrutement de médecins salariés. Une autre solution peut résider dans le soutien aux investissements nécessaires à la création de maisons de santé et de centres de santé, mais aussi dans l'expérimentation du recrutement de médecins salariés, en prévoyant une décharge des tâches de gestion administrative. Cette crise du médecin généraliste est une autre crise sanitaire qui touche les communes en plein coeur. Naturellement, en matière de désertification médicale, personne ne possède de baguette magique, et j'ai bien conscience que la réforme du portera ses fruits dans quelques années, mais il faut agir avant d'attendre. La situation de Cappelle-la-Grande est plus que parlante.

généralistes libéraux. La première évaluation du zonage montre que ces dispositifs incitatifs contribuent à freiner les difficultés démographiques régionales. Dans l'arrondissement de Dunkerque, 39 médecins

plus de 550 000 euros ont été mobilisés en ce sens. Les moyens sont donc là. L'autre levier renvoie à une meilleure organisation géographique des professionnels de santé, le développement des structures d'exercice coordonné,

À plus courte échéance, le Gouvernement a décidé la création de 4 000 postes d'assistants médicaux sur l'ensemble du territoire national, pour seconder et appuyer les médecins dans un ensemble de tâches administratives. Nous essayons donc de prendre

aussi flagrante qu'inacceptable. Si des avancées récentes figurent dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 concernant les professionnels relevant de l'assurance maladie, si 400 millions d'euros sont débloqués pour le secteur de l'aide à domicile,

voire entre les catégories de professionnels eux-mêmes au sein d'un établissement. Les exemples sont multiples et les situations rapportées par certains responsables de ces structures médico-sociales privées à but non

plus que l'autre ? Autre incohérence : sur les six instituts médico-éducatifs (IME) présents sur le département, tout le personnel, y compris les services généraux et les administratifs, de l'IME Édouard-Seguin, lequel relève de la fonction publique

Le Gouvernement considère-t-il que les professionnels des secteurs médico-social et social ne sont pas aussi essentiels que les soignants dans la prise en charge des personnes vulnérables ou en situation de handicap ? Ce secteur connaît pourtant déjà de grandes difficultés de recrutement, qui menacent la capacité de prise en charge

Monsieur le sénateur Patrice Joly, s'il est un gouvernement qui s'est attaqué à la revalorisation des professionnels du secteur médico-social, c'est bien le nôtre. Je n'avais pas entendu parler de prime covid pour les auxiliaires de vie ; nous l'avons fait. Je n'avais pas entendu parler de revalorisation pour le personnel des établissements

d'un complément de traitement indiciaire (CTI) pour les personnels des établissements de santé et des Ehpad. Cette mesure a été étendue par la signature de trois accords de méthode dans le cadre de la mission confiée à Michel Laforcade. Le Gouvernement a présenté devant chacune des deux chambres du Parlement des amendements à étendre le bénéfice de la mesure socle aux personnels soignants, aux auxiliaires de vie sociale, aux aides médico-psychologiques ou aux accompagnants éducatifs et sociaux exerçant dans des établissements et dans des services accompagnant des personnes handicapées et financés par les conseils départementaux, ainsi que dans les accueils de jours autonomes et dans les résidences autonomie. autonomie. L'ensemble de ces mesures avait vocation à entrer en vigueur dès le 1 novembre 2021 dans le secteur privé non lucratif, pour les personnels éligibles. Depuis cette date, l'ensemble des soignants

qui affectent le rendement des cultures, rompent l'équilibre de l'environnement qu'elles colonisent, et, surtout, dont le pollen est hautement allergène pour l'homme. Certes, des mesures réglementaires

de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2019 et à la publication du plan d'action pour la lutte contre les ambroisies dans ce département. Celui-ci précise les actions nécessaires à mettre en oeuvre, comme la surveillance des ambroisies et l'information du public à son sujet, ou encore l'entretien régulier des bords de routes et des cours d'eau. Toutefois, force est de constater que les résultats de ces initiatives demeurent très insuffisants, et l'inexorable invasion de l'ambroisie appelle aujourd'hui une mobilisation de plus grande envergure. Je souhaite donc vous interroger sur deux points. Premièrement, quels nouveaux moyens techniques le Gouvernement compte-t-il déployer pour agir beaucoup plus efficacement ? Deuxièmement, de quels instruments juridiques envisage-t-il de doter les collectivités territoriales pour leur permettre d'agir plus efficacement en faveur de la prévention et de la lutte contre l'ambroisie malgré leurs efforts soutenus, les communes resteront désarmées si elles ne bénéficient pas de nouvelles prérogatives, notamment coercitives, pour faire appliquer les mesures prises contre la propagation de cette plante. La parole est à Mme la ministre

a estimé, dans un récent rapport, qu'entre 1,1 et 3,5 millions de Français étaient allergiques à l'ambroisie. Selon ce rapport, le coût de leur prise en charge médicale est estimé à 59 millions d'euros, celui des arrêts de travail à 10 millions d'euros et celui des pertes de qualité de vie à 350 millions d'euros par an, au minimum. Afin d'organiser la prévention que vous évoquez, les préfets de département ont autorité pour arrêter les mesures visant à prévenir l'apparition de ces espèces ou à lutter contre leur prolifération en fonction du contexte local. Il s'agit, par exemple, d'organiser leur surveillance, ainsi que l'information du public et des acteurs concernés. L'obligation de destruction des espèces sous quelque forme que ce soit au cours de leur développement fait également partie des mesures de lutte inscrites arrêtés préfectoraux pris depuis 2017, notamment dans l'ensemble des départements de votre région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est fortement affectée. Le succès de la lutte contre l'ambroisie est un enjeu majeur, qui ne sera réglé que par la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes. Nous animons, notamment, cette lutte au travers du troisième plan régional santé environnement, l'agence régionale de santé (ARS), vise à réduire l'exposition de la population aux pollens allergisants en assurant la surveillance de l'exposition, en sensibilisant aux risques, en développant des outils de gestion et en promouvant des actions de lutte dédiées. Des innovations techniques voient le jour, notamment en matière de surveillance, par l'emploi de données satellites ou de drones. Des équipes de recherche travaillent à l'amélioration des connaissances pour mieux lutter, y compris au moyen de l'insecte, contre

Pour ces personnels, aujourd'hui, la durée maximale de travail est fixée à 48 heures par semaine. Si le code du travail permet de solliciter une dérogation à hauteur de 60 heures maximum, le code rural autorise, quant à lui, à demander une dérogation jusqu'à 72 heures.

Homogénéiser ou réduire ces heures n'est pourtant pas envisageable, en raison des contraintes climatiques et naturelles inhérentes à chaque forme de culture. Le monde agricole nécessite de tels aménagements. Le Gouvernement va-t-il soutenir le travail manuel et saisonnier ? La parole

notamment lors des vendanges, pendant lesquelles les besoins de main-d'oeuvre sont accrus. L'inspection du travail considère toutefois que les vendanges ne constituent pas, à elles seules, une circonstance exceptionnelle susceptible de justifier légalement le recours à la suspension du repos hebdomadaire. Cette position se justifie, puisque, si une dérogation est demandée chaque année, on ne peut logiquement plus arguer du caractère exceptionnel et imprévisible de la demande. voudrais toutefois vous rassurer : la réglementation en vigueur offre beaucoup de souplesse aux viticulteurs, afin de leur permettre d'adapter leur temps de travail au rythme des vendanges. le code rural et de la pêche maritime leur permet déjà de déroger au repos dominical. Ainsi, sur deux semaines, un viticulteur pourra être en mesure de travailler jusqu'à douze jours consécutifs, s'il prend son repos le lundi de la première semaine et le dimanche de la semaine suivante. Par ailleurs, les viticulteurs peuvent solliciter une dérogation aux durées maximales journalières et hebdomadaires ; la durée quotidienne peut être portée à 12 heures et la durée hebdomadaire à 60 heures, voire à 72 heures. Ainsi, notre droit permet bien à la filière viticole d'aménager la durée du travail au rythme des vendanges. Cependant, il n'est pas souhaitable, pour la santé d'un viticulteur, de suspendre le repos hebdomadaire après avoir travaillé dans les vignes 132 heures pendant douze jours consécutifs. C'est là une question de santé à laquelle nous ne pouvons déroger.

Faut-il rappeler que nous avons vécu une année marquée par des aléas climatiques d'une ampleur inédite ? Les moissons ont été particulièrement difficiles et se sont étalées dans le temps.

En 2019, il obtient son CAP, ainsi que la médaille d'argent départementale au concours du meilleur apprenti de France. Toutefois, ce parcours exemplaire est arrêté net en janvier 2020 par une notification d'obligation de quitter le territoire français Malheureusement, cet exemple n'est pas unique. De nombreux jeunes étrangers sont victimes de ce curieux mécanisme. Arrivés en France alors qu'ils sont mineurs et sans leur famille, ils sont pris en charge et s'inscrivent dans un parcours de formation pour mieux s'intégrer. Leurs efforts se voient étrangement récompensés ... Qu'ils soient inscrits dans un cursus d'apprentissage ou qu'ils soient en emploi, rien n'y fait. L'âge de la majorité atteint, le titre de séjour nécessaire à la poursuite de leur progression leur est refusé. Incompréhensible humainement, ce dispositif l'est tout autant du point de vue financier et économique. En effet, la France investit dans l'éducation de ces jeunes, pour ensuite leur interdire de poursuivre leur cheminement dans la vie active. Que dire, enfin, des conséquences néfastes subies par les entreprises qui les intègrent en alternance pour mieux les employer ensuite ? Orientés vers des secteurs professionnels en tension, ces jeunes migrants sont autant de forces vives qui manquent malheureusement à notre économie.

Afin de prévenir les ruptures de droit à la majorité et de sécuriser les parcours d'intégration des mineurs non accompagnés, il a été mis en place un examen anticipé du droit au séjour à la majorité, dès que les jeunes ont atteint l'âge de 16 ans ou 17 ans. Une instruction en ce sens a été signée et diffusée le 21 septembre 2020. Ainsi, lorsque le mineur se présente à la préfecture pour y solliciter une autorisation de travail dans le cadre de son insertion professionnelle, on lui propose que son droit au séjour soit examiné de manière anticipée. Dans un premier temps, donc bien en amont de la majorité, les vérifications portent sur les documents d'état civil, de nationalité et et de domicile. Si des difficultés sont détectées à ce stade, dans le cadre de l'expertise documentaire notamment, le mineur dispose de plusieurs mois, avec l'accompagnement du conseil départemental, pour solliciter les autorités consulaires compétentes. Dans un second temps sont vérifiées les autres conditions, notamment le suivi de la formation, la nature des liens avec le pays d'origine, le degré d'insertion de l'intéressé et l'absence de menace pour l'ordre public. À l'issue de cet examen en deux temps, le conseil départemental est informé par écrit des conclusions sur le droit au séjour du mineur étranger, permettant ainsi à ce dernier d'engager le cas échéant toutes les démarches nécessaires, afin de lever les difficultés. Par ailleurs, les services du ministère de l'intérieur ont adressé en février 2021 aux services des préfectures un état des lieux des bonnes pratiques à mettre en oeuvre,

été donnée. Le flou juridique qui entoure la disparition non inquiétante de majeurs responsables pose un frein important à la poursuite de recherches judiciaires, dans les quelque 40 000 à 50 000 cas de personnes disparues recensés chaque année. On estime parallèlement qu'environ 1 000 à 1 500 personnes sont enterrées anonymement durant la même période. Déjà évoquée auprès des services du ministère de l'intérieur par le passé, la constitution d'un fichier national d'empreintes permettrait d'identifier des dépouilles retrouvées et ainsi de les croiser avec des empreintes génétiques de personnes disparues. À l'heure actuelle, un simple prélèvement ADN pourrait en effet se révéler particulièrement concluant aux fins de clore définitivement des affaires restées non résolues, de sorte que les familles enfin se délester d'un deuil devenu impossible à accomplir. Une identification par voie dentaire serait intéressante à privilégier, compte tenu de la résistance et du caractère faiblement dégradable de l'émail dentaire, ainsi que de la densité d'informations génétiques contenues dans la dentition. Elle fait en outre déjà l'objet d'une application au sein de la cellule « Renseignement Famille » de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN). L'élargissement de ce dispositif aux personnes enterrées sous X, qui se matérialiserait sous la forme d'un projet déjà évoqué depuis 2018 sous le nom de Fenix, pour désigner le fichier d'enregistrement et d'identification des X, permettrait de réduire le faisceau d'incertitudes sur les personnes recherchées. La création de ce fichier semble toutefois dormir dans les placards du ministère ... Face au consensus des experts médicaux et dentaires et à la demande des familles de personnes disparues,

Mme la ministre déléguée. Monsieur le sénateur Lefèvre, plusieurs outils informatiques développés au sein du ministère de l'intérieur peuvent répondre aux besoins d'identification des personnes décédées et enterrées sous X. En premier lieu, le fichier des personnes recherchées est un outil généraliste, consacré à la recherche et à la surveillance des personnes. Sont inscrites dans ce fichier les personnes disparues dans des conditions inquiétantes, ainsi que les personnes décédées ou vivantes non identifiées. Le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), quant à lui, permet d'enregistrer les auteurs d'infractions, les empreintes des cadavres non identifiés et celles des personnes disparues. En complément, le fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg) enregistre les profils des auteurs d'infractions, des cadavres sous X et des personnes disparues. Le décret du 29 octobre 2021 étend les possibilités d'enregistrement des profils ADN. Il permettra, à terme, de mettre en oeuvre une interconnexion avec la base ADN d'Interpol. police et la gendarmerie nationales ont également développé des fichiers spécialisés dans la collecte des données et des informations relatives aux personnes disparues, d'une part, et aux personnes et cadavres découverts et non identifiés, d'autre part. Au sein de la police nationale, la direction centrale de la police judiciaire a développé un projet de fichier d'enregistrement et d'identification des X (Fenix). Une fois qu'il sera autorisé par le Conseil d'État, le fichier Fenix permettra d'effectuer des rapprochements entre des données nationales et internationales. Il facilitera la comparaison d'un dossier de découverte d'un cadavre non identifié ou de personne hospitalisée sous X avec l'ensemble des personnes disparues. Il aidera les services enquêteurs à s'orienter sur de nouvelles pistes de recherches, notamment lorsque le décès ou la disparition remonte à plusieurs années.

de la jeunesse et des sports. Madame la ministre, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées garantit le droit à tout enfant « présentant un handicap ou un trouble de la ou un trouble de la santé invalidant d'être inscrit dans une école en milieu ordinaire ». Les unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS) sont des dispositifs permettant la scolarisation d'élèves en situation de handicap au sein d'établissements scolaires En Seine-Maritime, la rentrée de septembre 2021 a été chaotique pour de nombreux élèves de collège bénéficiant de ces dispositifs. En effet, à Sotteville-lès-Rouen, Bacqueville-en-Caux, Auffay, Saint-Saëns, Dieppe ou encore Saint-Nicolas-d'Aliermont, pour ne citer que ces communes, plusieurs établissements n'avaient pas d'enseignants spécialisés en septembre, car ceux qui s'y trouvaient en poste, issus du premier degré, avaient été réaffectés dans des classes du cycle élémentaire. Faute de candidats issus du secondaire, des contractuels non formés ont alors été recrutés à la hâte Pôle emploi. Or ils ont été nombreux à démissionner par la suite, dépassés face à des enfants qui ont des troubles et handicaps spécifiques. Trois mois plus tard, la situation des élèves en situation de handicap accueillis dans des établissements ordinaires reste loin d'être optimale, puisque les classes ULIS, censées recevoir des effectifs de 12 élèves au maximum, voire 10 élèves dans certains cas, voient ce plafond largement dépassé pour pallier le manque d'enseignants. Cela va à l'encontre des recommandations, qui visent à aménager un accueil adapté et une prise en charge du handicap par des équipes spécialisées. Cette situation nuit directement à la qualité de l'accompagnement, lequel subit déjà les conséquences d'une politique de recrutement favorisant les contractuels au détriment des enseignants spécialisés. La scolarisation des élèves en situation de handicap devrait être une priorité. Aussi, madame la ministre, quelles mesures le Gouvernement entend-il mettre en oeuvre pour mettre fin à ces dysfonctionnements et donner à ces dispositifs essentiels les moyens nécessaires pour accueillir les enfants comme il se doit

Dans le souci de renforcer les démarches inclusives dans tous les degrés d'enseignement, il a été décidé, en Seine-Maritime, de proposer les postes de coordonnateur ULIS au collège et en lycée uniquement pour le mouvement des enseignants du second degré. En plus d'une implication toujours plus grande des enseignants de collège et de lycée dans les dispositifs d'inclusion, ce choix permet d'affecter prioritairement les professeurs des écoles spécialisés dans des dispositifs en école ou dans des unités d'enseignement des établissements médico-sociaux dont les postes pouvaient rester vacants à l'année. De surcroît, afin d'assurer une meilleure inclusion scolaire dans le second degré, l'académie a déployé un important plan de formation des personnels du second degré et promeut activement les métiers de l'inclusion scolaire et la formation au certificat d'aptitude professionnelle Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ne mène pas une politique visant à privilégier une forme de recrutement par rapport à une autre. Il peut arriver, cependant, que nous soyons amenés à recruter du personnel contractuel, afin notamment de répondre à certains à certains besoins locaux. Ces nouveaux recrutés bénéficient d'un soutien renforcé, grâce à des sessions de formation spécifiques, ainsi que d'un accompagnement individuel en classe et hors de De manière générale, l'académie a engagé une dynamique ambitieuse d'ouverture de dispositifs ULIS, afin de répondre aux besoins de scolarisation adaptée d'un nombre croissant d'élèves. Ainsi, en Seine-Maritime, ce ne sont pas moins de 18 nouvelles unités qui ont été créées à la rentrée 2021, dont 5 en collège et 8 en lycée,

Le choix de l'anglais a été effectué également pour des raisons pratiques et de reconnaissance la plus large auprès des États où la carte d'identité peut être utilisée comme document de voyage. En outre, l'anglais figure parmi les vingt-quatre langues officielles et de travail de l'Union européenne. Telles sont les considérations qui ont conduit le ministère de l'intérieur à choisir la langue anglaise comme seconde langue

n° 1972, adressée à M. le ministre de l'intérieur. Ma question porte sur les conditions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle des communes ayant subi des dommages provoqués par les effets de vents cycloniques. Le 19 juin 2021, les communes de Saint-Nicolas-de-Bourgueil et de Bourgueil ont été traversées par une tornade d'une puissance exceptionnelle. L'observatoire français Keraunos a enregistré des vents oscillant entre 175 kilomètres par heure et 220 kilomètres par heure. Si aucune victime n'est à déplorer, les dégâts matériels sont considérables. À Saint-Nicolas-de-Bourgueil, commune d'un peu moins de 1 200 habitants, le clocher de l'église et le toit de la salle des fêtes ont été détruits. Une centaine d'habitations a été touchée, sans compter les chais, hangars et dépendances. Les vignes et la forêt ont été dévastées. En juillet dernier, le ministre de l'intérieur a pourtant refusé de reconnaître à cet événement l'état de catastrophe naturelle. En effet, l'intensité anormale de l'agent naturel ne serait pas caractérisée.

À défaut d'une reconnaissance d'état de catastrophe naturelle, les dommages sont indemnisés au titre de la garantie tempête, grêle, neige prévue par les contrats d'assurance des biens. De nombreux dégâts, tels que ceux qui sont subis par les routes, ouvrages, réseaux électriques, vignes et forêts, sont exclus de toute indemnisation.

Gouvernement envisage-t-il de modifier les critères applicables, afin d'ouvrir le bénéfice de cette garantie aux communes de métropole victimes de vents cycloniques ? Par ailleurs, quelles mesures particulières prendra-t-il pour aider ces deux communes et leurs habitants à reconstruire leurs villes ? La parole est à Mme la ministre Monsieur le sénateur Babary, l'événement qui a frappé Saint-Nicolas-de-Bourgueil le 19 juin dernier ne constitue effectivement pas un épisode de vents cycloniques couvert par la garantie catastrophes naturelles au sens de l'article L. 122-7 du code des assurances. effet, les vents n'étaient pas associés à un cyclone tropical, et leurs vitesses n'ont pas atteint les seuils fixés par la loi, qui correspondent à des cyclones de catégorie 4 ou 5. raison pour laquelle la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle de Saint-Nicolas-de-Bourgueil a été rejetée. En revanche, les dégâts sur les biens assurés des particuliers, des entreprises et des collectivités causés par des vents violents et par la grêle sont couverts par leur contrat d'assurance au titre de la garantie tempête, grêle, neige La garantie tempête, rendue obligatoire dans l'ensemble des contrats d'assurance dommage par le législateur, permet aux sinistrés d'être indemnisés par leur assureur sans qu'une intervention préalable des pouvoirs publics soit nécessaire. Ces phénomènes, qualifiés d'« assurables », car ils peuvent se produire sur l'ensemble du territoire national, sont indemnisés exclusivement par les assureurs. L'État n'intervient donc pas dans le déclenchement de leur prise en charge. Les habitants de Saint-Nicolas-de-Bourgueil sinistrés par la tornade du 19 mai dernier sont donc indemnisés directement par leur assureur sur le fondement de la garantie L'État mobilise par ailleurs d'autres dispositifs d'aide au profit de certaines catégories de sinistrés, tels que le régime des calamités agricoles ou le dispositif de dotation de solidarité en faveur des collectivités territoriales. différents dispositifs, adaptés aux caractéristiques des phénomènes naturels et à la situation particulière de chaque catégorie de sinistrés, permettent une indemnisation efficace des victimes d'un événement météorologique intense.

Dans toutes ces communes, les moyens sont limités. Pourtant, leurs mairies incarnent souvent le dernier service public et, plus souvent encore, le maire et ses adjoints sont les seuls représentants de l'État identifiés. Dans chacune d'entre elles, jusqu'aux plus petits villages, les secrétaires de mairie sont donc des appuis essentiels. Fonctionnaires de catégorie A à C, ils remplissent toutes les missions administratives de la commune,

Vous le savez, les plus petites de nos communes ne peuvent se permettre de disposer d'un secrétaire de mairie à temps plein, de sorte que les salaires sont en réalité plus faibles encore, à moins que les communes aient pu s'organiser à plusieurs pour partager le poste.

La Fédération nationale des centres de gestion a également transmis ses propositions au ministère de la transformation et de la fonction publiques. En effet, la problématique liée au métier de secrétaire de mairie des petites collectivités recouvre des réalités multiples. Les différents questionnements des secrétaires de mairie, ces 20 000 agents qui accomplissent une mission de service public et de soutien aux élus indispensable au bon fonctionnement de nos petites communes et plus largement du service public de proximité en zone rurale, font l'objet de toute l'attention du Gouvernement.

Ces propositions recouvrent des domaines tels que les dispositifs statutaires, les conditions d'emploi, les missions, la formation, les parcours professionnels et la rémunération ou l'environnement de travail. mesures sont en cours d'expertise et devraient permettre d'identifier et de présenter prochainement les leviers permettant d'apporter des réponses adaptées à ces problématiques. Nous comptons ainsi renforcer l'attractivité de ces emplois. Ces propositions s'ajoutent à celles déjà identifiées par le ministère de la transformation et de la fonction publiques,

À Bobigny, ville préfecture du département, 37 % des habitants se trouvent sous le seuil de pauvreté, et 70 % d'entre eux vivent en quartier prioritaire des politiques de la ville. Malgré ces difficultés, la ville de Bobigny cherche à instaurer une dynamique urbaine, notamment par le biais de deux projets dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain. Ainsi, Bobigny porte un projet de requalification des logements de la cité de l'Abreuvoir, dans le quartier Édouard Vaillant. Réalisée par Émile Aillaud, la cité de l'Abreuvoir est reconnue « Architecture contemporaine remarquable Pour réaliser au mieux ce projet de requalification et pour donner des moyens financiers à hauteur des ambitions aux maîtres d'ouvrage, la ville a déposé une demande de majoration pour excellence auprès de l'Agence Ce projet a été réalisé en partenariat avec le ministère de la culture, qui en a souligné le caractère exemplaire. Sa qualité a également été soulignée par l'ANRU, notamment du fait de sa prise en compte de la dimension patrimoniale, ainsi qu'en raison de l'amélioration considérable des conditions de vie pour les habitants, grâce à un niveau de réhabilitation important, le tout dans une perspective durable, avec l'objectif d'une labellisation ÉcoQuartier. Malgré ces qualités, qui correspondent par ailleurs aux critères de l'ANRU, cette majoration pour excellence a été refusée. Madame la ministre, quels seraient donc les critères attendus pour obtenir cette majoration, afin que cette requalification des logements nécessaire aux Balbyniens et Balbyniennes puisse se réaliser dans les meilleures conditions possible ? La parole Gay, le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), a pu être relancé et entrer en phase opérationnelle, grâce à la détermination du Gouvernement, ainsi qu'à celle des collectivités territoriales, d'Action Logement et du mouvement HLM. et du mouvement HLM. Cette mobilisation collective a permis de doubler l'enveloppe financière en 2018, puis de la porter à 12 milliards d'euros après la décision du Premier ministre d'un nouvel abondement de 2 milliards d'euros, dont 200 millions d'euros de contribution supplémentaire de l'État, lors du comité interministériel des villes de janvier dernier. Ce nouvel abondement était nécessaire pour accélérer les mises en chantier, tirer les conséquences de la crise sanitaire et tenir compte du renouvellement des conseils municipaux lors des dernières élections. seulement de finaliser la programmation, qui concernera 450 quartiers et plus de 3 millions d'habitants, mais aussi d'amplifier les projets existants dans le cadre de clauses de revoyure.

L'opération de requalification de la cité de l'Abreuvoir bénéficie d'un niveau de financement élevé, notamment au regard de réhabilitations comparables soutenues par l'ANRU. Le bailleur social bénéficie déjà de deux majorations pour cette opération, l'une en raison de l'objectif de performance énergétique des logements, l'autre pour soutenabilité financière. La majoration pour excellence que vous évoquez n'est pas une gratification allouée sur une analyse de qualité. Elle est destinée à accompagner des surcoûts induits par les objectifs qualitatifs de l'opération. À ce titre, deux majorations ont déjà été accordées. L'avis du comité d'engagement prévoit une possibilité pour le bailleur de faire état de coûts plus élevés que les ratios prévisionnels qu'il a utilisés à ce stade, à l'issue des études de maîtrise d'oeuvre et sur la base des marchés de travaux, ... Il faut conclure, madame la ministre déléguée. ... et d'utiliser alors les marges d'ajustement des concours financiers entre les opérations qu'il porte pour ce projet. La

Depuis le 1 janvier 2021, plusieurs opérations portant sur l'isolation des murs ou le remplacement de chaudières sont soumises à des contrôles, afin de lutter contre les abus des entreprises frauduleuses. Ces contrôles consistent en une visite et un rapport d'un bureau de contrôle.

Le retour du train de nuit est donc une bonne nouvelle, mais il ne marque pas le retour à la normale. Plusieurs interrogations restent en suspens. Monsieur le ministre, quelles seront les conséquences des derniers travaux sur la ligne ? La SNCF a d'ores et déjà annoncé la suppression des circulations le 29 janvier et les 11, 12, 19 et 26 mars 2022, afin de finaliser les travaux d'aménagement. Des solutions de substitution ferroviaire seront-elles proposées aux usagers ?

connaissent des difficultés de recrutement. Ces difficultés sont d'autant plus complexes que ces entreprises présentent des performances économiques faibles, qui s'érodent depuis plusieurs années, et que les résultats attendus pour 2021 ne s'annoncent pas bons. Il semble aujourd'hui que plus de 10 000 postes doivent être pourvus sur l'ensemble du territoire.

En effet, depuis le mois de septembre dernier, les dysfonctionnements se multiplient, conduisant à un ras-le-bol généralisé et légitime des voyageurs, qui, en ce qui les concerne, s'acquittent du prix du billet et remplissent donc leurs obligations. Face à l'incapacité chronique de la SNCF de rendre la pareille, et après deux ultimatums qui n'ont malheureusement pas fait le conseil régional des Hauts-de-France, dont je suis également l'élu et qui prend ses responsabilités en matière d'investissement, n'a eu d'autre choix que de suspendre sa participation financière au fonctionnement des lignes. Cette position est assumée, à raison, par Xavier Bertrand- je le soutiens sans réserve -, alors que le plafond des pénalités pour la suppression des trains a été atteint dès le mois Certes, la SNCF a mis en place, trop tardivement, le mois dernier, un plan d'urgence. Mais force est de constater que ses effets sont très limités et que ce dernier peine à produire des résultats concrets. Monsieur le ministre chargé des transports, pour défendre la SNCF, vous répondrez que cette dernière a pris toutes les mesures adéquates, qu'elle a dû gérer des tensions sur les effectifs de contrôleurs et de conducteurs et sur le matériel, ou qu'elle a même dû faire face à une augmentation de faits externes comme les aléas climatiques ... Cela n'explique malheureusement pas cette faillite sur une telle durée. Ces difficultés ne sont pas des cas isolés. Elles surviennent à répétition et entament la confiance des Français envers la SNCF.

en matière de trains supprimés. Cette dynamique doit se poursuivre, grâce à un complément d'agents roulants, une homogénéisation du parc et une réindustrialisation de sa maintenance. La SNCF proposera également un plan de qualité et un travail précis sur neuf lignes, en s'engageant à baisser le taux de trains supprimés à 3 %, au lieu de 8,5 % observés actuellement. Elle a donné son accord de principe pour effectuer les remboursements des abonnements aux usagers. Un effort sera effectué pour améliorer la communication et l'information des usagers en cas de retard ou suppression, notamment grâce à l'application « assistant SNCF », qui permet d'informer les clients en temps réel. Je salue la reprise d'un dialogue constructif entre la SNCF et la région Hauts-de-France. Les élus régionaux suivront l'avancée de ces travaux engagés et seront amenés à prendre les décisions qui préserveront au mieux les intérêts des habitants de la région et du département de l'Oise. Une réunion est prévue pour faire le point sur l'ensemble de ces sujets le 18 janvier prochain. La parole

En effet, les mineurs entretenaient autrefois des vignes dont certains cépages ont été interdits en 1934 : le clinton, le jacquez, le noah, et l'isabelle. Toutefois, nous savons désormais que certains de ces cépages, dominants dans les Cévennes, ne contiennent pas plus de méthanol que d'autres. Nombreux sont les Français à être de plus en plus curieux de cépages anciens et nombreux sont les producteurs attachés à préserver ce patrimoine immatériel. Ces cépages, dès lors qu'ils sont bien cultivés et bien vinifiés, donnent des arômes typiques à un vin de plus en plus recherché. De plus, ils ne nécessitent quasiment pas de traitement, comparés à la viticulture traditionnelle.

L'adaptation des pratiques aux enjeux environnementaux et au changement climatique est une priorité pour la filière viticole, comme pour l'ensemble des filières agricoles. Dans le cas de la réforme de la politique agricole commune (PAC), la France a soutenu l'évolution proposée par la Commission européenne d'autoriser la production de vin sous appellation d'origine protégée (AOP) à partir de cépages issus de croisements avec. En effet, En effet, l'introduction de ces cépages dans les AOP constitue l'un des leviers pour répondre aux défis de l'adaptation du vignoble non seulement aux évolutions des conditions climatiques, mais aussi aux préoccupations relatives à l'usage des produits phytosanitaires. Ces cépages issus des recherches récentes

Danone a annoncé la transformation de son usine de lait de Villecomtal-sur-Arros dans le Gers en un site de production de boissons végétales, pour fabriquer notamment du lait d'avoine. En convertissant son unité de fabrication de yaourts à base de lait, Danone entraîne des ruptures de contrat avec 230 exploitations laitières dans les départements du Gers, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, des Landes, du Lot et des Pyrénées-Atlantiques.

Beaucoup sont endettés, certains sont vieillissants : il leur est difficile, à plus de 55 ans, d'envisager de nouvelles perspectives d'évolution pour leurs exploitations agricoles. En outre, il est fort à craindre que la transformation de cette usine aura des répercussions lourdes sur les emplois directs et indirects pour le territoire des Pyrénées-Atlantiques, comme pour les départements voisins.

intervient dans un contexte de réorientation stratégique du groupe, mais aussi d'optimisation de ses sites de collecte. Le ministre de l'agriculture est parfaitement conscient qu'une telle réorientation suscite des inquiétudes pour les 230 exploitations laitières laitières qui en dépendent, comme pour les employées de cette usine, même si, à ce jour, l'usine est maintenue, mais avec des activités différentes. Nous suivrons la situation avec rigueur, afin qu'aucun éleveur ne soit laissé au bord du chemin.

Ces évolutions passeront par un dialogue soutenu et transparent entre Danone, les éleveurs et les organisations représentatives, en lien étroit avec l'État. Certaines discussions ont été d'ailleurs engagées ces dernières semaines dans un esprit constructif. Nous veillerons à ce que le dialogue perdure et aboutisse à des solutions pérennes. Cette situation montre aussi une nouvelle fois combien nous devons agir pour préserver notre souveraineté alimentaire. Ne nous voilons pas la face : cette décision a également été prise face à la déprise laitière de ces zones, qui rend les outils industriels parfois difficiles à rentabiliser.

au carrefour de la Méditerranée. Notre pays est particulièrement engagé dans le processus de paix en Libye, lequel a permis la constitution d'un gouvernement d'unité nationale. Des élections seront organisées le 24 décembre. À cette occasion, Paris a rouvert son ambassade à Tripoli en mars. Toutefois, sa section consulaire demeure délocalisée à Tunis. Les entreprises libyennes, publiques et privées, sollicitent la technicité des entreprises françaises dans des secteurs aussi divers que l'aviation, l'énergie, la santé ou le traitement de l'eau et l'assainissement. Or, à ma connaissance, un partenaire libyen souhaitant un visa d'affaires pour la France doit aujourd'hui se rendre à Tunis, y laisser son passeport quinze jours, puis y retourner pour le récupérer. entendu, ces chefs d'entreprise préfèrent désormais passer par le consulat italien de Tripoli où ils obtiennent un visa en deux jours, privant la France d'opportunités. Ces lourdeurs administratives ne sont pas étrangères à la dégringolade de notre pays dans la liste des partenaires commerciaux de la Libye, Libye, de la troisième place en 2010 à la huitième aujourd'hui. Il semble donc opportun de réagir ! Notre pays regorge de belles entreprises qui pourraient participer à la reconstruction de la Libye, que nous appelons tous de nos voeux. Or la France perd des parts de marchés face à ses concurrents italiens, allemands, turcs ou chinois. quand le consulat, ou à tout le moins une section consulaire, rouvrira-t-il à Tripoli pour permettre à des partenariats commerciaux de se nouer ou de se renouer entre la France et la Libye ? La parole est à M. le ministre

consécutive aux affrontements armés. Depuis lors, les services consulaires ont été relocalisés à Tunis et au Caire. Le Président de République a émis le souhait très fort de rouvrir une emprise diplomatique ; c'est le cas depuis le 29 mars dernier.

Nous disposons désormais d'un dispositif de sécurité permettant la protection de l'ambassadrice et des agents qui effectuent des déplacements, dont ceux du service économique. Vous

Pourtant, la situation économique se révèle très défavorable aux collectivités qui vendent des matériaux recyclables. Par ailleurs, le faible nombre de centres de collecte dans certains territoires ruraux fragilise l'activité de recyclage des

Il a également abaissé de 8 % à 3 % les frais de gestion perçus par l'État sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour les cinq premières années au cours desquelles s'appliquera le mécanisme de la part incitative.

relance. Monsieur le ministre, je souhaiterais attirer votre attention sur les modalités de remboursement des voyageurs en cas de faillite d'une agence de voyages. La recrudescence actuelle de l'épidémie fait en effet craindre de nouveau des annulations de séjour. Lors de la première vague, l'ordonnance du 25 mars 2020 avait prévu divers assouplissements, afin de préserver la trésorerie de ces agences.

dans le cas où l'organisateur ou le détaillant fait l'objet d'une procédure de faillite, de quelles garanties légales de remboursement dispose le voyageur ? Le cas échéant, l'État s'engage-t-il à se substituer aux agences de voyages défaillantes, notamment si le délai de remboursement est anormalement long ?

La politique numérique du département repose sur trois piliers complémentaires : les infrastructures, les services, les usages et la médiation numérique- accompagnement des publics pour l'émancipation numérique et la résilience. Cette politique fait l'objet d'une nouvelle feuille de route, qui sera mise en oeuvre tout au long de la mandature.

outre, comme vous le savez, pour que les touristes viennent et reviennent, il faut leur proposer un accès numérique de qualité. C'est un prérequis de l'offre touristique actuelle, et le Puy-de-Dôme a besoin de fortifier son attractivité touristique et économique.

Monsieur le ministre chargé du tourisme, je souhaite attirer votre attention sur la mention d'origine des produits de la pêche dans les restaurants. Si la zone de pêche et le pays d'élevage sont toujours précisés dans les poissonneries, tel n'est pas le cas dans les restaurants, alors même que c'est obligatoire pour la viande depuis un décret du 17 décembre 2002. Pour les produits de la pêche, selon l'article L. 412-6 du code de la consommation, qui a été introduit par la loi du 20 juin 2016 pour l'économie bleue, cette indication est facultative. Alors que la consommation locale a été très largement promue par la loi du 22 août dernier portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est légitime que le consommateur puisse être informé de l'origine des aliments qu'il consomme. Est en jeu également la valorisation de l'activité de nos pêcheurs et poissonniers, qui suivent des traditions ancestrales. Les restaurateurs sont, quant à eux, fiers de pouvoir inscrire à leur carte des produits locaux de qualité.

Aujourd'hui, la même situation se reproduit. Le prix des carburants en Guyane s'établit à un niveau encore jamais atteint, de loin le plus élevé de tous les départements et régions d'outre-mer (DROM), supérieur à celui qui avait conduit à la révolte de 2008

Monsieur le ministre, les Guyanais ne peuvent et ne veulent plus subir de telles augmentations, alors même que 53 % d'entre eux vivent en deçà du seuil de pauvreté. Il faut réagir, monsieur le ministre, et vite ! Il est plus que temps de mettre en oeuvre une formule de calcul des prix juste et effectivement contrôlable, ce qui n'est pas le cas

en effet la gestion du recouvrement de la taxe d'aménagement des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) vers la direction générale des finances publiques (DGFiP) et, surtout, elle en modifie les modalités de paiement. Cette taxe, due par le propriétaire d'un bien immobilier qui dépose un permis de construire ou une déclaration préalable de travaux, porte sur les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments existants, ainsi que sur les travaux de changement d'affectation. Jusqu'à présent, son produit était reversé à la collectivité dès l'autorisation de construire. Or, la loi prévoit que, à compter du 1 janvier 2023, le fait générateur sera, non plus le permis de construire, mais le dépôt de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux

à feu. Au cours des neuf premiers mois de cette année, les tentatives d'homicide ont augmenté de 100 % en Martinique, rien qu'en zone de police, les violences sexuelles ont bondi de 40 % et les vols à main armée de 18 %. La Martinique enregistre ainsi, sur cette même période et uniquement en zone de police, 45 tentatives d'homicide et 9 homicides. Par ailleurs, 40 policiers ont été blessés, certains ont subi des tirs à balles réelles et 52 armes à feu ont été saisies par les forces de l'ordre. Il est important de noter que, depuis 2020, la hausse de la violence et des crimes a continué de s'accentuer, ainsi que la circulation des armes sur l'ensemble de ce territoire. L'enjeu est important. Il y va de la protection des enfants, de la quiétude de l'île et de son attractivité. Face à cette hausse alarmante des faits de délinquance, madame la ministre, quelles mesures ambitieuses le Gouvernement a-t-il prises ? Quels moyens matériels et humains a-t-il déployés pour endiguer la violence et la prolifération d'armes à feu sur l'île, notamment à la suite de la réunion de décembre 2019, où le Gouvernement a détaillé ses priorités pour lutter contre l'insécurité ? La parole

Agissant de concert avec les moyens spéciaux de la section aérienne de gendarmerie et les véhicules blindés à roues de gendarmerie, ils ont permis le rétablissement de la circulation et de l'ordre républicain. Les opérations conduites sur le terrain ont en outre permis le placement en garde à vue de 42 individus et le déferrement de la moitié d'entre eux. Pour lutter contre la prolifération des armes, le commandement de la gendarmerie de Martinique a mis en place un plan « armes », qui coordonne l'action des unités dans ce domaine, avec des résultats intéressants : les saisies sont en hausse de 53 % depuis 2019. Au titre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, tout est mis en oeuvre pour éradiquer ces trafics. L'antenne de l'Office anti-stupéfiants (Ofast) peut en particulier s'appuyer sur deux structures récemment créées : la cellule du renseignement opérationnel sur les stupéfiants (Cross) et une antenne du service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée Le commandement de la gendarmerie s'appuie en la matière sur ses unités de recherche, qui participent au « bureau de liaison stupéfiants » animé par l'Ofast et le parquet de Fort-de-France. Des réunions bimensuelles sont également organisées avec la Cross 972, avec une orientation très opérationnelle. Pour aller encore plus loin, la création au 1 janvier 2022, en Martinique comme dans le reste de l'outre-mer, d'une direction de police unique, la direction territoriale de la police nationale plaçant sous un commandement unifié l'ensemble des forces permettra à la police nationale, par une optimisation des moyens et des structures, d'améliorer l'efficacité de sa gouvernance territoriale et ses capacités opérationnelles sur le terrain.

Parmi elles, il y avait 7 femmes et 3 jeunes. Leur embarcation serait partie du Dunkerquois, peut-être de Loon-Plage, pour tenter de rejoindre l'Angleterre. Ils ont été secourus par les bénévoles de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Calais. le phénomène des « embarcations de fortune », ces marins sont en première ligne. Ils constatent avec tristesse l'augmentation des interventions auprès d'embarcations de migrants dans la Manche depuis des années. Sur la zone Gris-Nez, la SNSM dénombre 143 interventions par les stations de Berck-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer, Calais, Gravelines et Dunkerque depuis le début de l'année 2021. La très grande majorité concernait des migrants. Ces interventions exigent des pleins de gasoil, des centaines de couvertures et des vivres. Elles mobilisent souvent les bénévoles plusieurs heures, parfois des nuits entières. L'intensité de ces opérations de sauvetage et leur multiplication n'altèrent en rien l'engagement des sauveteurs bénévoles. Néanmoins, le désarroi de ces exilés les ébranle. Ils ne pensaient pas être appelés un jour pour récupérer des cadavres en mer. Lors d'opérations difficiles, ils craignent pour la sécurité de leur équipage. Leur matériel, qu'ils entretiennent eux-mêmes, est mis à rude épreuve. La SNSM est une association à but non lucratif reconnue d'utilité publique, financée à 80 % par des dons.

La SNSM est un organisme indispensable dans l'organisation du sauvetage en mer- je tiens ici à saluer l'ensemble de ses membres pour le travail extraordinaire qu'ils réalisent. À ce titre, l'État apporte à cette association d'utilité publique Tout d'abord, le Centre ressource d'aide psychologique en mer, le Crapem, créé en 2020, se tient à la disposition et à l'écoute des marins des stations SNSM en soutien psychologique. « Ensuite, sur le plan financier,

L'État porte également une attention particulière à la condition de bénévole et a permis, entre autres, la reconnaissance et la valorisation de leurs formations, ainsi que l'attribution du statut de pupille de la République aux enfants de sauveteurs décédés en opération de sauvetage- malheureusement, il y en Le phénomène migratoire que connaît la Manche mobilise particulièrement tous les moyens de l'État, mais aussi, comme vous l'avez souligné, la SNSM. Afin de préserver au mieux la mobilisation des bénévoles, et devant la recrudescence des traversées, le préfet maritime a donné la consigne de ne solliciter la SNSM que pour les cas de sauvetage avérés. Si le nombre d'opérations de ce type pour la SNSM n'excède pas 8 % de l'ensemble des moyens mobilisés, cela représente tout de même pour les bénévoles plus de 150 sorties, dans des conditions très difficiles. Les sauveteurs en mer le sont par vocation, mais ils n'en restent pas moins des bénévoles, et il est de notre responsabilité de les préserver devant la grandeur de leur tâche. « Les stations du Nord-Pas-de-Calais ont vu leur activité croître et leurs frais de fonctionnement augmenter. L'organisation nationale de la SNSM permet à chaque station qui nécessiterait un soutien financier particulier d'être accompagnée par le siège, et je me suis bien assurée du plein soutien de la SNSM à ces stations. » La parole

a le droit de choisir qui elle accueille sur son territoire. C'est le point central d'une politique migratoire. Aussi cette question, que je pose au nom de ma collègue Valérie Boyer, retenue en circonscription, concerne principalement les flux migratoires entre la France et l'Algérie. En 2019, plus de 15 800 Algériens ont été visés par une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Seulement 10 % de ces mesures ont été exécutées.

ou en Europe ? Quand les OQTF cesseront-elles de n'être que de simples « invitations à partir », soumises au bon vouloir du pays d'origine des ressortissants ? La question de la maîtrise de nos flux migratoires et de l'immigration illégale n'est pas anodine, car notre modèle de protection sociale et notre modèle républicain en dépendent. Que penser également de notre surpopulation carcérale, quand près d'un quart des détenus écroués en France est étranger ? Pouvons-nous admettre un seul instant que ce chiffre alarmant puisse être la conséquence, plus ou moins directe, d'une politique migratoire défaillante ? Sans volonté politique pleinement affirmée dans ce domaine, c'est à terme

« Ainsi, les Algériens continuent de représenter la première nationalité au titre de l'activité d'éloignement avec 22 957 interpellations réalisées depuis le début de l'année 2021, contre 14 955 en 2019, et 12 231 OQTF prononcées sans délai de départ, contre 9 466 pour l'année 2019. « Depuis la fermeture de ses frontières en mars 2020, l'Algérie a réduit très nettement sa coopération en matière de réadmission. de l'année 2021, seuls 33 Algériens ont fait l'objet d'un éloignement forcé, contre 1 650 pour l'année 2019. « Cette dégradation de la coopération a pu s'expliquer au début de l'année 2020 par le contexte exceptionnel de l'épidémie de covid, mais elle ne se justifie plus aujourd'hui. Désormais, nous disposons des moyens de mettre en place des protocoles sanitaires adaptés pour réaliser des éloignements en toute sécurité. Le contexte sanitaire ne peut pas dédouaner les pays de respecter leurs obligations internationales : tout État doit réadmettre ses ressortissants en situation irrégulière. C'est la raison pour laquelle le Président de la République a décidé de prendre un certain nombre de mesures en matière de coopération consulaire avec l'Algérie, pour laquelle le nombre de visas délivrés par nos consulats va diminuer de moitié. Ces mesures sont d'application immédiate, mais elles sont progressives et réversibles, si nécessaire. Concernant la procédure de déchéance de la nationalité française, neuf déchéances de nationalité ont été prononcées sur décision du Premier ministre entre 2017 et 2021

vous m'interrogez sur le fonctionnement de Parcoursup et sur les améliorations à engager pour renforcer, encore et toujours, l'information des lycéens, leur accompagnement dans la construction de leur projet d'orientation.

et, depuis 2018, des progrès considérables ont été réalisés grâce à la mobilisation de tous. Nous avons tout d'abord rendu accessibles sur Parcoursup toutes les formations conduisant à des diplômes reconnus par l'État, y compris par la voie de l'apprentissage. Aujourd'hui, plus de 19 500 formations sont répertoriées.

qu'ils ont été accompagnés et aidés dans leur projet d'orientation. Ils ne sont jamais laissés seuls dans ces démarches : pour chaque classe de terminale, deux professeurs principaux accompagnent les élèves dans la procédure, en plus des personnels spécialisés dans l'orientation. Dans le cadre de la réforme du lycée, du lycée, un temps dédié à l'orientation a été mis en place pour la première fois, au plus près des élèves, sous des formes variées. L'information sur les métiers s'organise également avec les régions, dont vous savez qu'elles disposent désormais de compétences dans ce champ.

ce travail d'accompagnement doit parfois être plus structurel. C'est pourquoi, au travers des « cordées de la réussite », qui rassemblent aujourd'hui 185 000 collégiens et lycéens, nous travaillons à stimuler leur ambition et à combattre l'autocensure.

La question des aides à la mobilité pour les personnes en situation de handicap est un sujet extrêmement sensible. Il est effectivement essentiel que chaque personne utilisatrice d'un fauteuil roulant puisse bénéficier d'un moyen adapté à sa situation et à ses besoins.

Ce projet semble remettre fortement en cause les questions essentielles relatives au libre choix des aides à la mobilité les plus adaptées à la situation singulière de chaque utilisateur, notamment par l'imposition de modalités d'acquisition pour certains véhicules pour personnes en situation de handicap et de délais de renouvellement, par des limitations de cumul d'acquisition, par les modalités de « restitution » des véhicules, par les impacts sur le parc et sur les innovations.

constater que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 ne fait apparaître aucune indication ni aucune programmation budgétaire relative à ces réformes, pourtant majeures, qui ne pourront certainement pas se mener à budget constant.

Permettez-moi en premier lieu de rappeler les difficultés majeures qui nous ont conduits à proposer cette réforme, très attendue : le frein financier, bien sûr, en raison de prix parfois exorbitants et non justifiés- ils sont parmi les plus élevés en Europe

L'axe principal de la réforme porte sur la révision de la nomenclature et des conditions tarifaires de prise en charge des fauteuils roulants. Le panier de soins actuellement couvert est obsolète et nécessite d'être révisé, comme vous le soulignez très justement. Le projet vise donc plusieurs objectifs. Le premier consiste à permettre un accès simplifié et plus rapide à des fauteuils roulants de qualité. Le deuxième, et je m'engage formellement sur cet objectif, consiste à garantir que chaque personne puisse bénéficier du fauteuil roulant le plus adapté à sa situation et à ses besoins, en respectant son libre choix. Cela passe par le renforcement des exigences sur le parcours de prescription, le développement d'essais systématiques en condition de vie réelle. C'est ce que nous faisons en déployant l'expérimentation d'équipes locales d'accompagnement aux aides techniques, plébiscitée par tous. faire évoluer la tarification pour réduire, voire supprimer le reste à charge, par un encadrement des prix et par une amélioration du remboursement de l'assurance maladie. Cette réforme, nous la menons dans un dialogue étroit avec les associations représentatives. J'ai moi-même eu l'occasion de réunir les administrations et l'association APF France handicap jeudi dernier, pour apporter des clarifications attendues sur le sujet du renouvellement du fauteuil, qui s'effectuera évidemment au regard de l'évolution de la pathologie et de l'état d'usure S'agissant du cumul d'acquisition, une personne pourra toujours bénéficier de plusieurs fauteuils si le besoin est identifié et objectivé par l'équipe médicale : fauteuil manuel et électrique, fauteuil adapté à une activité sportive, etc. Ce qui nous guide ici, je le répète, c'est bien de faire en sorte que nul n'ait à attendre plusieurs mois ou à demander le soutien financier de ses proches pour être autonome. C'est à la solidarité nationale de le garantir.

En effet, s'il convient d'agir sur les prix parfois prohibitifs des fauteuils, il n'en reste pas moins que le reste à charge financier pour certains modèles demeure extrêmement lourd pour le bénéficiaire. termes du décret, il y a fort à parier que nombre de personnes en situation de handicap vont devoir se résoudre à faire l'acquisition ou le renouvellement de leurs fauteuils en fonction de leurs possibilités financières, et non en fonction de leurs besoins, ce qui est grave et peut-être même aggravant pour leur handicap. handicapées, le Gouvernement entend-il persister dans la rédaction d'un tel décret ? Allez-vous défendre le libre choix dans l'accès aux aides à la mobilité pour les personnes handicapées ? Comment comptez-vous limiter le reste à charge pour les bénéficiaires ?

le recours à de multiples financeurs. La révision de la nomenclature et des conditions tarifaires de prise en charge des fauteuils roulants ne se déroule pas à huis clos, entre quelques hauts fonctionnaires qui ignorent les besoins des personnes. Je vous rassure, elle est menée en étroite association

à des fauteuils roulants de qualité et à assurer que chaque personne utilisatrice d'un fauteuil roulant puisse bénéficier du fauteuil roulant le plus adapté à sa situation et à ses besoins, en garantissant- je le dis haut et fort -le libre choix. Pour réussir, nous mobilisons tous les leviers. Il ne s'agit pas de réaliser une économie pour l'assurance maladie. La réforme que nous portons se traduira par des dépenses supplémentaires, puisque les remboursements seront plus élevés qu'aujourd'hui. Cette hausse de la prise en charge est couplée avec une négociation menée par l'État avec les fabricants sur les tarifs de ces fauteuils, à qualité identique. Il nous faut parvenir à un niveau de prix qui permette à la fois de préserver les marges, pour garantir l'innovation et la compétitivité, tout en ne créant pas de rente de situation. C'est un objectif que nous devons tous partager ici. Je tiens à vous rassurer, les personnes qui continuent à avoir un usage de leur fauteuil n'auront pas à le restituer en cas de nouvelle acquisition. Nous souhaitons cependant dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, inciter au réemploi des aides techniques non utilisées,

Laure Darcos, auteure de la question n° 1959, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. La Cour des comptes vient de publier son rapport sur les finances publiques locales, et le moins que l'on puisse dire est que les élus locaux doivent faire face à une situation très incertaine. En 2020, les collectivités territoriales ont été confrontées à une dégradation inédite de leur situation financière, qui s'est traduite par une diminution importante de leurs investissements. Cette année, elles ont dû absorber le choc de la réforme de la fiscalité locale consécutive à la suppression de la taxe d'habitation, mais aussi la réduction des impôts de production des entreprises. Tous les niveaux de collectivités ont vu leur panier fiscal modifié, avec pour conséquence un bouleversement du lien entre les contribuables et leur territoire. Au niveau des communes, seuls les propriétaires fonciers vont désormais contribuer au financement des services publics. intercommunale, les EPCI, s'est considérablement réduit, et les départements ont perdu tout pouvoir de taux sur leurs ressources. Les régions, quant à elles, ne disposent plus de ressources tirées de l'activité économique locale. Le remplacement d'impôts locaux par l'attribution d'une fraction de TVA n'est pas de nature à réjouir les élus, notamment en Essonne, d'autant que, avec cette réforme, vous exposez plus sévèrement le panier fiscal des collectivités territoriales aux variations de la conjoncture économique. Si l'objectif d'alléger la charge pesant sur les entreprises et les ménages est louable, rien en revanche n'a été fait pour rationaliser la fiscalité locale, la simplifier et la rendre plus lisible. Dans ce contexte, madame la secrétaire sera la suivante : bien qu'il lui reste peu de temps pour agir, le Gouvernement entend-il s'engager clairement à conforter l'autonomie financière des collectivités territoriales et à définir des ressources fiscales adaptées à chacune d'entre elles ?

vous remercie de votre question, car elle lui permet de redire que l'État a été présent de façon constante aux côtés des collectivités pendant la crise. Elle voudrait toutefois tempérer votre analyse sur la dégradation de la situation financière du bloc communal. L'épargne brute a certes diminué de 5,5 % en 2020 par rapport à 2019, mais elle reste à un niveau élevé de 18 milliards d'euros, qui est supérieur à celui de 2018. Les premiers éléments d'exécution sur 2021 montrent un redressement très net de la situation, qui pourrait même revenir à un niveau meilleur que celui de 2019. en place un filet de sécurité garantissant à chaque commune et intercommunalité que ses ressources fiscales et domaniales en 2020 ne seraient pas inférieures à la moyenne de celles perçues entre 2017 et 2019, sans quoi l'État leur versera une dotation égale à la différence. Plus de 4 200 bénéficiaires ont reçu 185 millions d'euros au titre de 2020. Le dispositif a été reconduit en 2021 pour les recettes fiscales. En deuxième lieu, les autorités organisatrices de la mobilité ont bénéficié d'une avance remboursable égale à 8 % de leurs versements mobilité et à 35 % de leurs recettes tarifaires de 2019. ou AOM, ont ainsi bénéficié d'un montant total d'avances remboursables de 620 millions d'euros. En troisième lieu, l'État a remboursé aux collectivités la moitié du coût des achats de masques. Ce dispositif a bénéficié à 16 500 collectivités, pour 230 millions d'euros. En quatrième lieu, l'État a ouvert une dotation de 200 millions d'euros pour compenser une partie des pertes de recettes, notamment tarifaires, liées à l'exploitation en 2020 d'un service public industriel, commercial ou administratif. Plus de 2 900 communes et groupements devraient bénéficier du dispositif avant la fin de l'année 2021. Ce mécanisme est reconduit en 2021.

pérenne et dynamique, et que, d'autre part, les communes et les EPCI conservent plusieurs pouvoirs de taux et d'assiette sur des impôts locaux, comme la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ainsi qu'un pouvoir de tarifs sur plusieurs taxes sectorielles, comme la publicité ou le tourisme. La parole

Je souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés juridiques rencontrées par certains exploitants agricoles à la retraite. En effet, lorsque ceux-ci ont mis fin à leur activité professionnelle et ont fait valoir leur droit à la retraite, ils ont naturellement perdu leur statut d'exploitant agricole. Cette perte a eu pour conséquence qu'ils ne peuvent plus légalement conduire leur tracteur, puisqu'ils n'ont pas de permis B. B. L'alinéa 2 de l'article L. 221-2 du code de la route dispose que « les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière [ ...] sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils pendant la durée de leur activité agricole ou forestière sans être titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré dès lors qu'ils sont âgés d'au moins seize ans, sauf exceptions prévues par décret en Conseil d'État Or la loi ne prévoit rien concernant l'hypothèse selon laquelle, bien qu'ils soient retraités, ils auraient encore ponctuellement besoin de conduire un tracteur, notamment dans la sphère familiale. Vous n'êtes pas

est à Mme la secrétaire d'État. En effet, monsieur le sénateur, les réglementations françaises et européennes en matière de conduite de véhicules automobiles prévoient que le conducteur doit être en possession d'un permis de conduire dont la catégorie est définie à l'article R. 221-4 du code de la route. Cet article dispose que la catégorie de permis de conduire exigé pour la conduite d'un engin agricole ou forestier, à savoir B, BE, C1, C1E, C ou CE, est définie en fonction du poids total autorisé en charge du véhicule, auquel s'ajoute celui de sa remorque éventuelle. Par exception à cette disposition, comme vous l'avez signalé, l'alinéa 2 de l'article L. 221-2 du code de la route précise que « les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils pendant la durée de leur activité agricole ou forestière sans être titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré dès lors qu'ils sont âgés d'au moins seize ans, sauf exceptions prévues par décret en Conseil d'État ». Si l'engin agricole est rattaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole son conducteur, dès lors qu'il est âgé de plus de 16 ans, n'est pas tenu d'être titulaire du permis de conduire. Dans ces conditions, un retraité agricole conserve la possibilité de conduire un tracteur sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie B,